sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2021

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, avec un solde déficitaire de 49 milliards d'euros en 2020 et un déficit prévu de 27 milliards d'euros en 2021, les dépenses de la branche maladie explosent. Si vous aviez effectué des réformes structurelles pour préparer l'avenir, « prévoir pour anticiper » constituant l'essence même de l'action de tout gouvernement, nous pourrions tolérer un déficit de cette ampleur ; seulement là, ce n'est pas le cas. La forte diminution des recettes est due à un ralentissement économique majeur engendré par un confinement aussi forcé qu'économiquement suicidaire. Nous sommes le pays européen qui impose les mesures les plus drastiques et les plus incohérentes à l'encontre de ses entreprises. Un exemple les fleuristes pourront, ce vendredi, vendre des sapins en extérieur, pendant que les foires aux santons, toutes en extérieur elles aussi, sont interdites. Ou comment rayer de la carte quatre cents emplois, mais aussi une profession, une passion, une culture, une identité Si nous voulons redresser les comptes sociaux, il va falloir retrouver la raison et la liberté de travailler pour tous les commerçants, les artisans et les indépendants. D'autres conséquences dramatiques, humaines celles-là, sont annoncées. Santé publique France a publié un rapport qui indique : « La santé mentale des Français s'est significativement dégradée entre fin septembre et début novembre, avec une augmentation importante des états dépressifs pour l'ensemble de la population. » Car ce n'est plus un Président qui nous dirige, mais le Premier Soviet entouré d'un contrôlant chaque pan de notre vie quotidienne. Vladimir Emmanuelovitch Macron nous impose l'heure de sortie et l'heure de retour à notre domicile, avec qui et où nous pouvons nous déplacer, qui a le droit de travailler, qui a économiquement le droit de vivre ou de mourir, ce que nous pouvons consommer, ce que nous devons penser, ce que nous pouvons exprimer et même où nous devons prier. Et tout cela, en s'étant affranchi du devoir démocratique de rendre compte devant le Parlement Incapable de contrôler l'épidémie, votre gouvernement a décidé de contrôler le peuple. La République soviétique française est « en marche » ! Je rappelle Je rappelle que j'ai proposé deux pistes pour améliorer la situation financière et sanitaire. J'ai ainsi déposé une proposition de loi visant à verser le montant des amendes du confinement aux hôpitaux- cela représente au moins 165 millions d'euros. J'ai aussi cosigné une proposition de loi visant à indiquer le lieu de fabrication des médicaments et de leurs principes actifs sur leur conditionnement et notice. Il faut une transparence dans l'information et il faut soutenir la réorientation des dépenses de santé vers des médicaments français. Il en va de notre souveraineté, et donc de notre sécurité sanitaire. En trois ans, la Macronie a fabriqué un million de pauvres supplémentaires, soit dix millions au total, et cent mille sans domicile fixe de plus ! Le voilà, le nouveau monde antisocial d'Emmanuel Macron, car tout ne peut pas être mis sur le dos du pangolin. Il faut conclure ! Pour répondre à cette France en souffrance, il est temps de rétablir une véritable politique de solidarité et de justice sociale, en appliquant la priorité nationale à l'embauche, en tordant le bras à la Commission de Bruxelles,

a entrepris l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021 en responsabilité. Cette position l'a conduite à approuver certains des choix opérés par le Gouvernement et à s'opposer fermement à d'autres, tout en alertant sur ceux qui devront être faits demain, mais ne sont pas pour autant présents dans ce texte. C'est en responsabilité que le Sénat a accepté des tableaux d'équilibre aux déficits historiques et un endettement record, considérant que l'urgence du moment est de tout faire pour éviter l'effondrement de notre économie et de répondre par la solidarité nationale à ceux que la crise prive de leur emploi ou revenu. C'est en responsabilité que le Sénat a mené une « opération vérité » sur les charges respectives de l'État et de la sécurité sociale. À la sécurité sociale, les effets de la conjoncture sur les recettes et les dépenses de l'hôpital ; à l'État, la reprise de la dette hospitalière, les dépenses de Santé publique France et les compensations des mesures de compétitivité ou de pouvoir d'achat. Ce débat n'est ni théorique ni le fruit d'une vision corporatiste de la sécurité sociale. S'il faut un jour augmenter les cotisations, agir sur le niveau des prestations ou rembourser la dette, il faut que ce soit l'équilibre des assurances sociales qui le commande, et non la charge des transferts du budget de l'État. Dans le même esprit, le Sénat a alerté sur les années à venir. Nous sommes comme anesthésiés par une mobilisation massive d'argent public, mais le réveil sera douloureux et nous n'avons pas souhaité l'occulter. Il faudra redresser la barre, certes pas aujourd'hui, ni même peut-être demain, mais certainement dès après-demain, en tout cas le plus tôt possible pour l'avenir même de la protection sociale et la préservation de cet acquis si précieux dans la crise. Cela implique certes une réponse massive, mais pas forcément de laisser toutes les vannes ouvertes. La commission n'a pas toujours été audible sur ce point, mais elle maintient sa position et ne manquera pas de la rappeler le moment venu. encore en responsabilité que nous avons accepté la réforme de l'accès précoce aux médicaments ou la pérennisation des maisons de naissance, mais aussi fait part de nos interrogations sur l'allongement du congé de paternité et de nos questionnements, sinon de nos doutes, sur la capacité du Gouvernement à donner corps à ce projet porteur d'espoirs qu'est la nouvelle branche autonomie. Prenons garde aux promesses non tenues qui alimentent une défiance déjà très forte chez nos concitoyens De la même manière, la fraude aux prestations comme aux cotisations sape les fondements de notre contrat social et, à l'initiative du rapporteur général de notre commission, le Sénat a substantiellement enrichi le volet fraude de ce projet de loi. La nécessité d'une réforme des retraites devant l'évolution de notre démographie s'était imposée avant la crise ; elle demeure d'actualité. La crise n'a pas fait disparaître ce problème, elle n'a fait que l'amplifier. Nous verrons si le Gouvernement mais aussi tous ceux à qui la position de la commission a fait pousser des cris d'orfraie ne sont pas contraints d'y revenir ... Je rappelle que le texte transmis au Sénat sur le système universel de retraite n'a pas été retiré certains membres du Gouvernement ont rappelé l'actualité de cette réforme. Il faudra bien la mener un jour. Nous ne pouvons pas non plus tarder sur la réforme du système de santé, dont la crise a certes montré les forces et l'excellence, mais aussi les rigidités et les cloisonnements. L'innovation est coûteuse ; elle nous invite à revoir les organisations, à révolutionner les parcours, ou elle remettra en cause un modèle solidaire auquel nous sommes tous ici profondément attachés. Il y a bien un modèle social « à la française » qui n'a pas fait défaut pendant la crise et continue à soutenir les malades, les retraités et les plus précaires. Pour qu'il continue de le faire demain, des réformes sont nécessaires. C'est le discours que la commission a souhaité porter. Animé de cette même conviction, le groupe Les Républicains votera ce texte. La parole La parole est à Mme Colette Mélot, pour le groupe Les Indépendants- République et Territoires.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons examiné la semaine dernière le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Les débats ont été l'occasion de dresser un premier état des lieux de notre système de santé,

Nous la devons aussi à toutes les victimes collatérales de la crise sanitaire, les commerçants, les restaurateurs, les artisans, les artistes et tant d'autres dans de multiples secteurs qui font face aux répercussions économiques et sociales des mesures sanitaires. Des mesures graves mais nécessaires, qui appellent un financement exceptionnel, limité aux quelques années à venir. Aussi, le texte que nous avons examiné comporte un certain nombre de mesures d'urgence, mais n'élude pas la question de réformes plus structurelles, issues notamment du Ségur de la santé.

d'assurance maladie (OCAM) sera mise en place au titre des années 2020 et 2021, sachant que le Sénat a adopté une mesure de différenciation des taux applicables selon le caractère lucratif ou non de l'organisme visé. Alors que la crise sanitaire a provoqué une forte augmentation des dépenses de la branche maladie, les organismes complémentaires ont économisé 2 milliards d'euros de remboursement durant la crise. Aussi, il nous semble que cette contribution est justifiée. D'autres mesures conjoncturelles importantes ont été adaptées à l'évolution de la crise et votées. Il s'agit de la prolongation du dispositif d'indemnité en cas d'activité partielle et de la création d'un dispositif complémentaire d'exonération des bénéfices pour les secteurs fermés totalement ou situés dans les zones de couvre-feu et ayant subi une baisse d'activité. À l'initiative du Gouvernement, les conditions de baisse d'activité ont été assouplies pour les secteurs dépendants des secteurs les plus affectés. Il s'agit d'une mesure très attendue par de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur culturel. La concrétisation des conclusions du Ségur de la santé constitue l'une des principales avancées du PLFSS pour 2021. Au premier rang figure la revalorisation des salaires des personnels soignants, paramédicaux et non médicaux à l'hôpital et en Ehpad. Ces mesures sont essentielles pour améliorer l'attractivité des métiers du soin et du secteur médico-social. Nous saluons également l'adoption d'une enveloppe de 200 millions d'euros dédiée au secteur de l'aide à domicile, qui sera versée aux départements par la Caisse Le Sénat a adopté plusieurs amendements visant à rationaliser le dispositif proposé par le Gouvernement. Nous saluons aussi la dotation du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé de 6 milliards d'euros, dont le champ des bénéficiaires a été étendu aux cabinets libéraux. En réponse au problème de l'engorgement des urgences, le texte prévoit la mise en place d'un forfait payant de 18 euros en remplacement du forfait de réorientation jamais appliqué. Nous sommes sceptiques sur l'efficacité d'un tel dispositif qui pourrait se traduire par un renoncement aux soins et une aggravation de l'état de santé des patients les plus précaires. Néanmoins, nous saluons l'adoption des mesures d'exonération de ce forfait, notamment pour les personnes souffrant d'une affection de longue durée Le Sénat a également adopté un nouveau dispositif, défendu par notre groupe, permettant à titre expérimental le développement de l'offre de téléconsultation en amont du passage aux urgences dans les établissements de santé. Je voudrais saluer la création d'une dotation finançant une mission d'intérêt général dédiée à la prise en charge des femmes victimes de violences. Hier, le ministère de l'intérieur a rendu un premier bilan à la suite du Grenelle des violences conjugales, indiquant une hausse de 16 % du nombre de victimes en 2019. Plusieurs dispositions visent à favoriser l'accessibilité des soins sur l'ensemble du territoire. Je pense notamment à l'amendement adopté par le Sénat qui vise à encourager la poursuite d'activité des professionnels de santé situés dans les déserts médicaux qui choisissent de continuer à exercer au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. L'instauration d'une durée légale minimale de quatre mois de stockage pour les médicaments à intérêt thérapeutique majeur va également contribuer à renforcer la continuité des soins, notamment pour les malades du cancer. Le texte prévoit des mesures importantes concernant la politique familiale. Nous saluons ainsi l'adoption du doublement du congé de paternité. Les amendements visant à assouplir cette mesure ont tous été repoussés. Nous savons qu'il existe de fortes disparités de prise de ce congé selon le type de contrat de travail. Le versement de la prime de naissance a été avancé avant la fin du mois civil suivant le sixième mois de grossesse. C'est une mesure très attendue qui permettra aux familles de mieux préparer l'accueil de l'enfant. Enfin, nous sommes bien sûr favorables à la généralisation des maisons de naissance qui seront aussi des lieux de prévention, d'éducation thérapeutique et de formation pour les sages-femmes. Nous saluons les avancées adoptées en matière de prise en charge de la dépendance et d'adaptation de la société au vieillissement de la population, mais nous restons dans l'expectative de la loi sur le grand âge et sur le financement de la cinquième branche, sachant que plus de 6 milliards d'euros sont attendus pour couvrir les besoins. Le Sénat a fait le choix de supprimer la reprise des 13 milliards d'euros de dette hospitalière par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades), Nous avons des réserves au sujet des dispositions relatives à la réforme des retraites. Si nous sommes favorables sur le fond au recul progressif de l'âge d'ouverture des droits à 63 ans, il ne nous paraît pas opportun d'introduire dans le contexte actuel au détour d'un amendement. Forts de ce constat partagé, une large majorité de notre groupe s'abstiendra et certains d'entre nous voteront en faveur de ce projet de loi.

après cette première lecture au Sénat, non seulement le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 n'a bénéficié que de peu d'amendements répondant aux défis sanitaires et sociaux, mais il repart lesté d'amendements régressifs. Il nous a fallu défendre les quelques avancées que nous avions saluées, comme l'allongement du congé de paternité, et qui sous couvert de considérations économiques ont fait l'objet de tentatives pour en contraindre l'accès. Alors que nous devrions consacrer l'essentiel de nos débats à construire la protection sociale de notre temps et à proposer les pistes de financement la rendant possible, ce projet de loi a moins que jamais suivi ce cheminement logique, seul susceptible de ne pas faire du PLFSS un outil d'austérité. Comme d'habitude, le Gouvernement détermine l'enveloppe fermée des ressources et refuse toutes les propositions pour en desserrer l'étau par une taxation plus juste des revenus et des patrimoines. La crise économique n'a que trop focalisé nos débats sur la politique d'exonération des cotisations sociales- celle-ci n'a rien de nouveau, mais elle connaît dans ce contexte une explosion inédite. Si l'intervention de l'État en soutien de l'économie est nécessaire- elle devrait cependant être modulée, conditionnée, et exclure de l'aide ceux qui profitent du contexte pour licencier -, nous regrettons que n'aient pas été au centre de nos débats la crise sociale et les mesures sociales à prendre immédiatement pour contrer le basculement dans la pauvreté, le chômage, la précarité et la dégradation de l'état de santé de la population. À chaque proposition de mesures sociales nouvelles, nos amendements sont déclarés irrecevables puisqu'ils entraînent des dépenses, et lorsque nous proposons de nouvelles ressources, celles-ci sont rejetées pour des raisons dogmatiques. Pour le Gouvernement et la majorité du Sénat, il n'est donc pas d'actualité, par exemple, de réintégrer pour les oubliés du Ségur les revalorisations ou les primes covid. Ces travailleurs sociaux et médico-sociaux- assistants familiaux et bien d'autres -qui ont contribué, en première ligne, à répondre à la crise sanitaire resteront donc des invisibles. Il n'est pas plus d'actualité de rechercher des ressources supplémentaires pour financer la cinquième branche, ou mettre fin à la destruction de l'hôpital public et à la marchandisation des champs du social et du médico-social, facteur de croissance des inégalités. Nous pouvons certes acter l'adoption de quelques amendements : la différenciation des taxes selon le statut des organismes complémentaires, même si nous récusons l'augmentation de leur fiscalité une mesure destinée à lutter contre le non-recours aux prestations par les personnes en situation de précarité sociale ; ou encore le rétablissement de l'opposabilité des accords de la branche du domicile garantissant l'égalité territoriale. Nous nous félicitons aussi de la suppression du transfert vers la sécurité sociale du financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), ainsi que de la suppression de la surcotisation salariale des sapeurs-pompiers. La crise sanitaire inédite que nous traversons rend encore plus inacceptable l'absence de volonté politique de récupérer les milliards d'euros de l'évasion fiscale,

Tous les amendements pour y remédier ont été rejetés, les nôtres comme ceux d'autres groupes que nous avons soutenus. comment combler ce déficit de ressources qui, face à des prestations dynamiques et à la création d'une nouvelle branche, fabrique le fameux trou de la sécurité sociale ?

tous les partenaires sociaux refusent la réouverture inopportune, voire indécente, de ce dossier au vu des urgences immédiates de la crise actuelle alors même que ce projet est contesté par une majorité de Français et d'organisations syndicales. Alors que la France enregistre des centaines de milliers de nouveaux chômeurs et que la moitié des retraités ne sont plus dans l'emploi au moment de la liquidation de leur retraite, la majorité sénatoriale n'a rien de plus urgent à proposer que de reculer l'âge de la retraite, véritable obsession idéologique.

à 2021 ! Permettez-moi tout de même de rappeler la position des écologistes sur le projet gouvernemental de réforme des retraites, lequel répond si bien aux attentes de la droite que celle-ci en demande la mise en oeuvre rapide, rapide, passant outre l'échec probable et annoncé d'une conférence de financement avec les partenaires sociaux. Cette contre-réforme vise à transformer profondément la logique solidaire, à unifier par le bas, à livrer ce risque aux produits de retraite par capitalisation de grands groupes à l'affût de ce qui n'est, pour eux, qu'un marché lucratif. Les écologistes défendent le système par répartition et par annuité, militent pour la réduction du temps de travail, y compris sur l'ensemble de la carrière, s'opposent aux allongements successifs de l'âge légal de départ à la retraite et pour le bénéfice du taux plein. proposent une prise en compte inédite de la pénibilité des activités en vue de réduire les années d'écart d'espérance de vie en bonne santé entre catégories socioprofessionnelles- je rappelle que cet écart est de presque dix ans entre un ouvrier et un cadre.

la contribution des revenus du capital, qui demeure l'une

Monsieur le président, madame la ministre, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour nos concitoyens touchés par le virus et leurs familles, ainsi que pour les salariés et les entreprises des secteurs les plus exposés. une pensée, enfin, pour les deux millions de professionnels de santé mobilisés, alors que notre pays est frappé par la deuxième vague d'une épidémie mondiale. L'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale est toujours un exercice particulier. Il l'est d'autant plus aujourd'hui qu'une crise sanitaire sans précédent a bouleversé nos sociétés. Ce PLFSS devait être exceptionnel ; il l'est à bien des égards. Il est exceptionnel par les moyens qui sont mis en oeuvre pour lutter contre l'épidémie, en soutenant la modernisation de nos hôpitaux et les personnels soignants. Grâce à ce texte, ce sont 1,8 million de professionnels et, parmi eux, l'ensemble des personnels paramédicaux des hôpitaux et des Ehpad qui bénéficieront d'une revalorisation salariale inédite et tant attendue. La traduction des accords du Ségur de la santé constitue ainsi une avancée majeure et les 19 milliards d'euros dédiés à l'investissement permettront de s'assurer de s'assurer que notre système de soins devienne plus efficient et plus moderne. Il est exceptionnel, aussi, par l'ambition des mesures sociétales qu'il permet de concrétiser. nous nous félicitons de l'adoption de certaines dispositions essentielles, en particulier l'allongement du congé de paternité de quatorze à vingt-huit jours, dont sept jours obligatoires. Cette réforme historique répond à une demande de la société de mieux impliquer le deuxième parent dans l'éducation des enfants et de rééquilibrer les tâches familiales dès la naissance. Par cette disposition, et malgré des débats parfois vifs, notamment sur le caractère obligatoire du congé, nous mettons en oeuvre, mes chers collègues, un outil efficace pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous nous en réjouissons ce texte répond également aux besoins des familles adoptantes, en allongeant le congé de dix à seize semaines. La pérennisation des maisons de naissance est une autre belle concrétisation de ce projet de loi et donnera aux sages-femmes les possibilités nouvelles qu'elles méritent. De même, l'adoption de l'amendement, porté par notre groupe, visant à s'assurer de la juste mise en oeuvre de la peine de privation de la pension de réversion ou de veuf pour les conjoints survivants coupables de violences conjugales, est une avancée essentielle. La lutte contre ces violences se doit d'être menée en profondeur et nous nous félicitons que ces mesures soient prises dès à présent. Enfin, nos débats ont aussi dessiné les prémices d'un nouvel engagement. Je pense à celui qu'a pris M. le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, concernant le remboursement des capteurs de glycémie pour les enfants de moins de quatre ans insulinodépendants et insulinorequérants. En permettant la mise en oeuvre de la cinquième branche dédiée à l'autonomie, le PLFSS concrétise enfin une avancée majeure. Nous entendons les critiques qui ont pu être émises sur son financement ou sa gouvernance, mais les faits sont là, mes chers collègues : promesse de longue date maintes fois repoussée par les gouvernements successifs, cette nouvelle branche dédiée au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap était réclamée depuis vingt ans. C'est d'ailleurs, rappelons-le, la première fois qu'est créée une nouvelle branche depuis 1945. La CNSA, qui sera chargée de la gestion de cette cinquième branche, sera dotée de recettes propres, ce qui permettra justement de répondre aux espoirs et aux attentes légitimes qu'elle suscite. Le soutien accru aux secteurs les plus touchés par la crise sanitaire est un élément central de ce PLFSS. Je pense en particulier au tourisme, à la restauration, au sport, à la culture et à l'événementiel, dont l'activité est fortement réduite, pour ne pas dire inexistante, depuis plus de huit mois. L'introduction d'un dispositif complémentaire d'exonération au bénéfice des entreprises des secteurs dits « S1 » apparaît également essentielle au regard des difficultés que rencontrent un certain nombre d'entreprises et, à travers elles, des millions de salariés. Ce texte, par les avancées multiples qu'il concrétise, répond donc à la gravité de la situation, mais les débats au sein de notre assemblée ont aussi mis en lumière un certain nombre de désaccords sincères. Je pense notamment à la suppression de l'expérimentation sur la pratique des IVG instrumentales par les sages-femmes, qui permettrait de pallier le manque de médecins pratiquant l'avortement, en particulier dans les territoires ruraux. Cela constitue un recul non négligeable. De plus, l'encadrement de la reprise partielle de la dette des établissements de santé assurant le service public hospitalier répond à un devoir de solidarité, en permettant à ces établissements de santé publics d'investir. La suppression de cette disposition en séance publique nous paraît aller à l'encontre de la nécessité de les accompagner en favorisant la pérennité de leur financement. Enfin, alors que nous débattions des mesures concrètes visant à lutter contre l'épidémie, sauver notre système de santé et soutenir les secteurs les plus touchés, la majorité sénatoriale a fait le choix de cliver sur une mesure controversée. Je veux redire, au nom du groupe RDPI, notre opposition à l'amendement adopté par la majorité sénatoriale visant, notamment, à repousser l'âge de départ à la retraite à 63 ans. Nous nous y opposons tant sur la forme que sur le fond. Nous regrettons la volonté de la majorité sénatoriale de profiter de cette crise sanitaire pour imposer aux Français une réforme paramétrique des retraites, laquelle aurait nécessité une large concertation associant l'ensemble des partenaires sociaux. Nous nous interrogeons également sur le moment choisi pour faire une telle proposition, discutable sur le fond, alors que notre pays traverse une crise économique et sociale sans précédent, qui bouleverse notre quotidien et frappe un grand nombre de secteurs. Les discussions sont d'ailleurs toujours en cours entre le Gouvernement et les partenaires sociaux. Il est donc particulièrement inopportun de vouloir accélérer le rythme d'une réforme profonde, qui nécessite du temps. nous regrettons ces mesures, tant la période que nous vivons implique, selon nous, un devoir de responsabilité afin d'apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par nos soignants, nos TPE, nos PME, nos indépendants et notre jeunesse, laquelle, nous le savons, lutte pour entrer sur le marché de l'emploi aujourd'hui encore plus qu'hier. Pour conclure, je dirai que, en dépit des nombreuses avancées que comporte ce texte, les modifications apportées par la majorité sénatoriale suscitent plusieurs désaccords importants. L'année 2020 restera exceptionnelle la question des retraites, remise chaque année sur la table par la majorité sénatoriale, n'avait aucunement sa place au sein de ce PLFSS 2021 ambitieux, examiné en période de crise. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI s'abstiendra sur ce texte. La parole

! Telle est la conséquence naturelle d'une chute spectaculaire des recettes et d'une augmentation tout aussi spectaculaire des dépenses. Oui, la pandémie et ses multiples conséquences ont durablement aggravé les comptes de la sécurité sociale, lesquels connaissaient une embellie depuis quelques années. Mais des choix ont été faits pour tenter de préserver la santé de nos concitoyens et de nos entreprises, des mesures qui étaient nécessaires. En ce sens, il s'agit aussi d'un PLFSS de responsabilité. Malgré le contexte, ce PLFSS de crise ne renonce pas à tout et fait émerger de bonnes mesures, par lesquelles j'aimerais entamer mon propos. il prévoit 8,8 milliards d'euros pour la revalorisation des salaires, avec notamment une augmentation visée de 15 % pour les aides à domicile, et de 183 euros par mois pour les personnels hospitaliers et des Ehpad. Ce rattrapage était attendu. Ensuite, il contient une avancée sociale majeure qui a fait débat au sein de notre hémicycle, avant d'être adoptée à la quasi-unanimité : l'allongement du congé paternité. La vision patriarcale de la société a vécu. Les pères ne veulent plus être traités comme des parents de seconde zone. Aujourd'hui, l'arrivée d'un enfant est un événement qui bouleverse l'existence des deux parents, qui cherchent ensemble à construire une parentalité fondée sur la proximité affective. Je ne reviendrai pas sur les nombreux bienfaits de cette mesure sur le développement de l'enfant. Je rappellerai seulement qu'il s'agit d'une véritable avancée pour l'égalité entre les femmes et les hommes, avancée très attendue par les jeunes générations. Nous

à faire des maisons de naissance des lieux de formation et de prévention, et à les déployer sur le territoire. Nous saluons, par ailleurs, l'accord trouvé avec le Gouvernement sur le soutien aux entreprises touchées par le couvre-feu et le reconfinement, en particulier celles qui dépendent de secteurs directement touchés. Attaché à la défense de la ruralité et des terroirs, le groupe RDSE se félicite aussi des mesures de soutien apportées au secteur agricole, notamment au bénéfice des travailleurs occasionnels et des jeunes agriculteurs. de l'allégement des cotisations sociales pour les non-salariés de la culture de la vigne ayant subi des pertes de chiffre d'affaires, combat porté par ma collègue Nathalie Delattre. Concernant l'organisation de notre système de santé, il me faut évoquer l'adoption d'un amendement, que nous avons été nombreux ici à porter, prévoyant de réduire d'un an le report de la convention médicale actuelle entre l'assurance maladie et les médecins libéraux. Nous avons beaucoup parlé de l'hôpital, alors que les appels à remettre les généralistes au coeur du système se multiplient, à juste titre : les liens ville-hôpital sont les garants du bon fonctionnement de notre système de soins. Nos médecins libéraux sont nos personnels personnels de premier recours, mais ils se sentent aujourd'hui oubliés. Repousser trop loin les négociations conventionnelles sur leurs conditions de travail et de tarification ne serait pas un bon signal. Les mesures de transparence adoptées par le Sénat vont aussi dans le sens d'une avancée, avec notamment une plus grande lisibilité demandée aux agences régionales de santé (ARS) sur l'utilisation des deniers publics et l'allocation des ressources financières aux activités de santé. Enfin, je souligne une autre mesure d'importance sur un sujet que le Sénat porte depuis plusieurs années : l'instauration d'un stock minimal de quatre mois pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Les pénuries de médicaments et de vaccins s'intensifient et mettent en danger la santé de nos concitoyens. La question de la responsabilité de l'État et des laboratoires ne doit pas être occultée. Ce sont des actes que nous attendons, et je me réjouis que le Sénat tienne ferme ses positions.

plus le maintien du forfait patient urgences (FPU) qui, sans être assorti de mesures en amont, ne remplira jamais son rôle de désengorgement des urgences et ne fera qu'accroître le reste à charge des patients ou le renoncement aux soins, nous ne soutiendrons les dispositions votées par la majorité sénatoriale au sujet des retraites. Certes, il existe un problème structurel, nous partageons ce constat. Mais dans cet hémicycle où nous prônons sur toutes les travées, les bienfaits de la concertation, il nous semble important de défendre, pour une réforme d'une telle ampleur, un débat et un véhicule législatifs à la hauteur de l'enjeu. dirai que ce PLFSS voit émerger de bonnes mesures et quelques marqueurs pour l'avenir, telle la création de la cinquième branche autonomie, même si son financement reste encore à préciser. d'une part, l'État persiste à ne pas compenser certaines charges indûment confiées à la sécurité sociale, contrairement à l'esprit de la loi Veil de 1994. D'autre part, l'augmentation de l'Ondam est cette année conjoncturelle, et vise à répondre à la crise. Permettez-moi de rappeler, madame la ministre, que des changements majeurs sont attendus, notamment depuis le Ségur de la santé. Aucun texte n'y a, pour l'heure, répondu. Espérons donc que, dans les prochains mois, une nouvelle réforme d'organisation du système de santé verra le jour pour concrétiser, conformément aux engagements du Gouvernement, les attentes fortes des Français, des professionnels et des élus. Cette organisation doit laisser davantage de place à la proximité, à la décentralisation et à la souplesse pour les acteurs de terrain. Espérons aussi qu'elle ne subisse pas le sort des réformes des retraites et du grand âge, trop de fois reportées.

L'absence, jusqu'au bout, du ministre de la santé n'est pas pour nous apaiser ! Déception et colère, car ce PLFSS n'est pas à la hauteur de la crise que nous affrontons et de ce qu'elle a révélé. Il ne résout aucun des problèmes soulevés par les personnels soignants et non soignants des secteurs de la santé et du médico-social. Vous qualifiez d'extraordinaire ce PLFSS, madame la ministre, parce qu'il débloque les 8 milliards d'euros du Ségur de la santé et 4 milliards d'euros pour la covid-19. Mais vous oubliez de dire que c'est conjoncturel, et que vous avez prévu de « serrer les boulons » dès la crise passée. Vous avez refusé, comme la majorité de droite du Sénat, de faire entrer de nouvelles recettes taxant le capital, qui profite de la crise. Les grands groupes du CAC 40 peuvent dormir sur leurs deux oreilles, notamment Sanofi, laboratoire pharmaceutique parmi les leaders européens qui va pouvoir continuer à fermer ses sites de recherche et de production en France et licencier à tour de bras, tout en versant des dividendes indécents à ses actionnaires ! Aucune intervention de l'État n'est envisagée pour avoir la maîtrise publique de la production et de la distribution des médicaments, alors que la crise de la covid-19 a révélé plus fortement que jamais une pénurie de médicaments, et que vous refusez de constituer des stocks suffisants. Quant aux mesures censées renforcer notre système de santé, pallier les difficultés et les manques criants de personnel, de matériel, de locaux, elles vont à l'encontre de l'intérêt commun. Au lieu d'ouvrir des lits d'amont et d'aval, vous imposez un forfait à 18 euros pour, soi-disant, lutter contre la saturation des urgences, ce qui est une absurdité économique et pose un grave problème de santé publique. Au lieu d'oeuvrer pour un meilleur maillage de l'offre de soins dans les communes, vous portez un coup grave aux centres de santé, en exigeant un conventionnement sélectif par les ARS pour toute nouvelle ouverture dans les zones surdotées. C'est un obstacle supplémentaire pour les centres de santé. d'une méconnaissance totale des valeurs qui les fondent, après l'introduction il y a deux ans de la possibilité pour les libéraux d'y exercer leur activité Face aux départs de plus en plus nombreux de professionnels de santé, aucun plan de formation et de recrutement n'est envisagé. Inutile, dès lors, d'espérer une amélioration de leurs conditions de travail. Pourtant, chacune et chacun, ici, a rendu hommage aux médecins, aux infirmières et infirmiers, aux aides-soignantes et aides-soignants, aux brancardiers. Mais quelle traduction réelle dans ce PLFSS ? Alors que la psychiatrie et la pédopsychiatrie sont sinistrées, ce PLFSS n'ouvre même pas sur une grande loi de santé mentale et poursuit une réforme tarifaire à base de tarification pas davantage de mesures significatives pour mettre en oeuvre le fameux « tester, tracer, isoler ». Et aucune prise en charge à 100 % pour les masques, devenus obligatoires dès l'âge

est un rendez-vous manqué, malgré quelques mesures positives que nous avons soutenues, comme l'allongement du congé paternité- mais nous en avons souligné les limites. Rendez-vous manqué, madame la ministre, car le gouvernement auquel vous appartenez reste sur les mêmes orientations politiques qui ont conduit notre système de santé là où il en est aujourd'hui. Vous refusez d'investir dans le système de santé pour ne pas augmenter la dette transmise aux futures générations. Mais si l'investissement consiste à construire des hôpitaux, des Ehpad, des centres médico-psychologiques (CMP), les futures générations seront bien contentes d'avoir cette créance pour leur prise en charge, dans un contexte de vieillissement de la population ce refus de suivre une autre voie, le jour d'après, avec vous, sera pire que le jour d'avant ! Cette voie conduit notre système de santé dans le mur, et pas seulement l'hôpital, car rien n'est prévu non plus pour la médecine de ville face au manque cruel de généralistes, et rien sur la mise à contribution des établissements privés pour la prise en charge des malades de la covid-19. Hélas, quoique mortifère, cette voie est également suivie par la majorité de droite du Sénat qui a aggravé les mesures régressives de ce PLFSS en votant, en pleine crise de la covid, le recul de l'âge de départ à la retraite à 63 ans et l'allongement de la durée de cotisations à 43 annuités. Ce sont les faits, totalement indécent, au moment où les plans de licenciement explosent et où de nombreux jeunes en recherche d'un travail vont devoir pointer à Pôle emploi. Le prétexte du comblement du déficit de la caisse des retraites ne tient pas, car il se double d'un refus d'envisager d'autres recettes. recettes. Pour l'ensemble des membres de notre groupe, ce PLFSS, c'est non ! Non à un budget insuffisant ! Non à un budget décalé de la réalité de la crise sanitaire ! Non au manque de reconnaissance des professionnels des secteurs de la santé et du médico-social Non à l'absence de plan de formation et de recrutements ! Non, enfin, au refus de mise à contribution des plus riches et des dividendes ! Nous disons, au groupe communiste républicain citoyen et écologiste, qu'un budget de la sécurité sociale pour 2021 tenant compte

sans capital. La seule qui ne va pas dans la poche des actionnaires mais est directement investie pour le bien-être de nos citoyens. Faire appel au budget des contribuables pour la financer serait subordonner l'efficacité de la politique sociale à des considérations purement financières. Ce que nous refusons. » Le groupe CRCE le refuse

Est-ce le manque de sommeil, l'intensité parfois des échanges, la valse des milliards, l'incongruité à vouloir prévoir l'avenir budgétaire, alors que personne ne sait où nous allons ? Ou encore les innovations, souvent importantes, introduites par ce texte, et quelques inévitables déceptions ?

appelait des mesures d'ajustement budgétaire afin d'amortir, autant que faire se peut, le surcoût engendré par l'épidémie de covid, et les dispositions du Ségur de la santé. Ainsi, le fait marquant de ce PLFSS est sans aucun doute cet abyssal déficit de 49 milliards d'euros de premiers secours. À situation exceptionnelle, remèdes exceptionnels ! Ainsi, chronologiquement fut d'abord votée une contribution des organismes complémentaires en santé. La modulation pour les organismes mutualistes a entraîné, dès la première heure, un manque à gagner de 400 millions d'euros. J'ai alors songé que, dans nos collectivités territoriales, on ne votait pas une mesure sans connaître son impact budgétaire. Il serait bon que les parlementaires disposent systématiquement des mêmes outils d'appréciation. C'était une remarque préliminaire L'un des objets de ce PLFSS était de permettre la mise en oeuvre des mesures du Ségur de la santé, en particulier l'augmentation salariale des personnels des établissements de santé et des Ehpad, et le financement de la prime exceptionnelle pour les personnels des services d'aide à domicile. Je veux dire un mot, ici, pour tous ceux qui se sentent oubliés du Ségur, exclus de la reconnaissance nationale.

La santé est un système vaste et complexe qui va bien au-delà des murs de l'hôpital, et les applaudissements symboliques des Français sont allés, dans les moments les plus durs, à chacun des acteurs de cette longue chaîne humaine. Dans la suite de nos débats, l'article 6 a marqué la volonté forte du Gouvernement d'aider les employeurs par une exonération totale de contributions sociales. Cela illustre le « quoi qu'il en coûte » qui, dans les heures de grand doute et de désespoir, doit être une planche de salut. Le champ de cette mesure est large. Espérons seulement qu'il n'y ait pas trop de trous dans la raquette ... Merci, madame la ministre, de mettre en oeuvre ces véritables outils de solidarité nationale. Je note l'adoption, aux articles 13 et suivants, de l'exonération des cotisations sociales pour les salariés non agricoles des exploitations viticoles, ainsi que la pérennisation et le relèvement du taux du dispositif d'exonération pour les travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, dits « TO-DE ». Espérant pour ces filières que ces mesures puissent prospérer, je souligne ainsi un exemple concret de soutien aux professionnels. Puis vint le moment de créer cette fameuse « cinquième branche », cette décision de traiter à part entière la dépendance, de donner un cadre aux futures mesures du grand âge et de la perte d'autonomie. De nombreuses questions et inquiétudes subsistent sur son financement, qui ne pourra pas reposer principalement sur la contribution sociale généralisée (CSG), son périmètre et sa gouvernance. Était-ce le moment ? Le rapport Libault prévoyait cette création à l'occasion de l'extinction de la dette sociale, afin que puisse être utilisé le produit de la CRDS pour soutenir cette branche.

Notre collègue Jocelyne Guidez, par ses remarques sur l'AEEH, nous invite par ailleurs à nous interroger sur la portée symbolique des dispositions. Un individu porteur d'un handicap est-il d'abord porteur de handicap, ou d'abord un enfant ? Puis, porteur de handicap ou retraité ? C'est la difficulté de classer les êtres humains dans des cases ... Ce texte apporte des avancées attendues et des propositions innovantes- versement anticipé de la prime de naissance ; création des maisons de naissance ; hôtels hospitaliers -, ainsi que cette mesure fort médiatisée visant à allonger le congé de paternité à vingt-huit jours, dont sept obligatoires. Me singularisant un peu dans cet hémicycle, j'ai exprimé ma crainte que l'on aggrave ainsi le fossé existant dans notre société entre ceux qui ont un salaire et ceux qui n'en ont pas. le Sénat, dans son immense majorité et sa très grande sagesse, a franchi ce pas. Médicaments innovants, stocks, téléconsultation, pénurie de professionnels de santé, répartition territoriale des médecins, dette hospitalière, médecine hospitalière, médecine de ville, médecine privée, sport et santé, périnatalité, concertation sur l'âge de la retraite ... tout le champ des sujets d'une brûlante acuité dans ce contexte sanitaire a été longuement balayé.

Notre collègue Nathalie Goulet a déposé de nombreux amendements relatifs à ce problème car elle maîtrise parfaitement ce dossier, qui est par ailleurs pointé dans nombre de rapports publics et officiels. Alors que le simple croisement de fichiers permettrait de mettre fin à bien des pratiques malhonnêtes, on se demande si l'atonie des débats ne confirme pas une forme de banalisation de la fraude. Madame la ministre, devant tous ces amendements qui ont été déclarés « satisfaits je réponds que nous ne sommes pas satisfaits ! Pour lutter contre la fraude, il faut plus que des lois, il faut une volonté ! Beaucoup de mesures relèvent du réglementaire, à vous de les prendre ! Plus que jamais, en période d'austérité et de rigueur, les Français vous attendent sur ce sujet.

Je vous donne un exemple : les préparations magistrales de mélatonine, qui permettent aux enfants autistes de trouver le sommeil, ne sont pas remboursées par la sécurité sociale.

Je rejoins ceux de mes collègues qui ont appelé à une refonte profonde et concertée de notre système de santé. Je conclus en remerciant ceux qui nous ont accompagnés pendant de longues heures,

écrire une loi de financement de la sécurité sociale conforme à la réalité dans ses équilibres financiers est une gageure, alors que nul ne sait précisément ce que le coronavirus, qui a déjà coûté la vie à 45 000 de nos compatriotes, nous réserve pour 2021. La question n'est évidemment pas de se prononcer sur cette adéquation : ce PLFSS établira probablement un record d'imprécisions. C'est plus que jamais le sens politique du texte qui engage notre avis. Voilà huit jours, à cette même tribune, je dressais le constat d'un rendez-vous manqué. Au sortir de son examen par notre assemblée, quelques dispositifs intéressants utiles plus tard, mais aussi après quelques reculs voulus souvent par la majorité de notre assemblée, le constat reste le même. Le rendez-vous avec l'hôpital reste inachevé, partiel et conjoncturel. Rien ne change dans la gouvernance et trop peu dans les moyens. Les urgences sont encore et toujours abordées sous le seul angle d'un dispositif de nature financière. Les soignants de ville, eux, restent destinataires de discours inappliqués sur leur rôle essentiel. Les aides à domicile devront se contenter de bien peu. Quant à la démocratie sanitaire, tellement malmenée depuis le printemps, oubliée jusqu'à compromettre l'adhésion de la population aux mesures de lutte contre l'épidémie, elle continuera à être marginalisée. Et si l'ajout de 100 millions d'euros déconcentrés vers les ARS doit être salué, rien dans votre amendement ne nous dit si la logique de leur engagement sera encore une fois purement verticale, ou si les acteurs des territoires Comme toute loi de financement de la sécurité sociale, celle-ci comporte des points positifs qui méritent d'être relevés. C'est le cas du congé paternité et de la création de maisons de naissance, par exemple. J'ajouterai plusieurs mesures qu'a proposées, ou auxquelles a contribué, notre groupe : la lutte contre le non-recours aux aides sociales ; la pérennisation du dispositif TO-DE ; l'obligation de constitution d'un stock de quatre mois pour les médicaments majeurs, alors que tant de malades sont victimes de ces ruptures le renforcement de la protection des patients soumis à des mesures de contrainte en psychiatrie ; le retour de l'Agence nationale de santé publique dans le budget de l'État. Cela ne dissipe pas notre inquiétude face à votre choix de « charger la barque » du budget social dans son exécution annuelle et dans son endettement, lequel s'accroît de ce qui devrait être à la charge du budget de l'État. Les conditions mêmes d'examen du texte disent beaucoup. Présenté très tardivement, dépourvu d'étude d'impact sur des dispositions introduites, elles aussi, tardivement, examiné en moins de temps qu'il n'en faut pour que le travail soit suffisamment approfondi, il a de plus été modifié significativement par le Gouvernement en cours de

La conférence des financeurs est certes un outil nécessaire, mais sans la visibilité qu'offrirait une nouvelle loi relative au grand âge et à l'autonomie, que pourra-t-elle décider ? Le temps des crises doit être celui des changements. Cette crise n'est pas un accident de l'histoire. En son lendemain, il ne suffira pas de reprendre une trajectoire de rétablissement des comptes sociaux, comme certains discours le laissent entendre. Cette crise est systémique et doit nous amener à revoir notre système de santé et à repenser le sens de notre protection sociale. Elle a d'ores et déjà révélé des défauts organisationnels majeurs de l'État et de notre gouvernance en matière de santé publique, ainsi qu'une crise de la décision.

L'État central a présenté des failles inquiétantes et la part nécessaire de décentralisation de notre politique de santé est absente de ce texte. Ce n'est d'ailleurs pas surprenant, puisque le ministre de la santé, qui ne nous fait toujours pas l'honneur d'être présent a exprimé son opposition à cette orientation. L'amendement n° 201 porte un privilège rare : à lui seul, il disqualifie le texte qui nous est proposé.

leur demandent de travailler plus longtemps. Ils le demandent même aux plus pauvres, pour des pensions qui seront inévitablement plus faibles, et ce alors que la majorité sénatoriale refuse avec constance- je le regrette ! -l'idée d'une contribution des plus riches à la situation exceptionnelle que nous vivons. C'est votre choix, que vous avez fait devant la Nation par votre vote. Mais pour nous, c'est non ! Ce budget social est un budget d'injustice sociale ! Ce n'est pas acceptable, et nous l'exprimerons par un vote négatif sur ce texte. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

résultat du scrutin. Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques

Le travail parlementaire se poursuivra, puisque vous allez vous réunir avec vos collègues députés en commission mixte paritaire. Sans préjuger de l'issue de celle-ci, je tiens à saluer quelques avancées majeures que vous avez introduites ou entérinées. Dans le contexte sanitaire actuel, que chacun a rappelé, je pense en premier lieu au relèvement de 800 millions d'euros de l'Ondam, en plus des 2,4 milliards d'euros déjà votés par l'Assemblée nationale. Ce relèvement permet de financer la stratégie de tests de la population, ainsi que les surcoûts induits par les outils de protection supplémentaire des professionnels dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Je salue également le soutien que vous avez apporté à l'allongement du congé de paternité,

et que les départements n'y contribueront pas, alors que c'est de leur compétence et que nous y travaillons déjà ensemble. Je suis persuadée que, par le dialogue avec l'ensemble des parlementaires des deux chambres, nous parviendrons à un équilibre. Je suis très attachée à ce dialogue et j'espère que nous pourrons le poursuivre en bonne intelligence. Les Français l'attendent. Nous serons, ensemble, à la hauteur du moment ! Mes chers

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire sans précédent que nous connaissons a mis en lumière, parmi les sujets que nous pensions- funeste erreur ! -acquis, celui de l'alimentation, celui de notre alimentation.

Oui, cette crise nous rappelle toute l'importance de ce que nous pouvons nommer la « sécurité alimentaire », le besoin de savoir que l'on pourra s'alimenter en quantité mais aussi en qualité suffisantes

Oui, monsieur le ministre, nous sommes nombreux, sur ces travées et dans nos territoires, à penser qu'il est désormais urgent de donner à l'alimentation un véritable statut. Il est temps d'en faire définitivement un secteur d'activité d'importance vitale, tel que défini par l'article R. 1332-2 du code de la défense, plutôt que de continuer de s'en tenir à sa seule dimension sanitaire.

Concept de la saisonnalité, enfin, avec la redécouverte de produits locaux et de saison, et une palette de productions qui permet de mélanger allégrement les goûts et les couleurs. Ce constat posé, quelles pistes explorer pour faire en sorte que le monde d'après ne ressemble pas au monde d'avant, et pour que ce moment éphémère, dont certains producteurs nous disent qu'il n'est déjà plus qu'un vague souvenir pour des consommateurs qui ont retrouvé leurs habitudes antérieures, donne le top départ d'une résilience alimentaire partagée par toutes et tous ? Derrière cela, c'est toute la question de notre souveraineté alimentaire qui ressurgit. Je sais, monsieur le ministre, que vous en avez fait la priorité des priorités. « Nous ne pouvons plus déléguer notre alimentation », indiquait le 12 mars dernier le Président de la République. La France est un grand pays agricole exportateur, mais elle est aussi un pays qui s'est inspiré du modèle américain mondialisé. Or ce modèle nous fait transférer d'énormes flux d'intrants, d'énergie ou d'azote du Brésil, pour nourrir des animaux que nous exportons ensuite vers le Moyen-Orient,

Au risque d'enfoncer des portes ouvertes, il nous faut réaffirmer un principe fort : reconstituer nombre de filières qui ne peuvent être que maraîchères, ou presque, le sud de la France étant, par exemple, fort touché par le changement climatique. Alors que nous exportons des volailles, nous importons 40 % des poulets que nous mangeons ; il convient de corriger cette inadéquation pour que la relocalisation de qualité prenne tout son sens. Pour les viandes, nous importons principalement les produits les moins chers, souvent pour la restauration collective. Sécurité alimentaire, souveraineté alimentaire, garantie d'un accès à une alimentation de qualité pour nos concitoyens, notamment pour celles et ceux qui subissent le plus la précarité, préservation de la biodiversité voilà, monsieur le ministre, les piliers qui devraient inspirer des contrats alimentaires territoriaux passés avec les collectivités, véritables feuilles de route pour une transition agricole et alimentaire partagée par le plus grand nombre.

Ils auront aussi pour vocation d'édicter des principes forts en matière de gestion du foncier agricole, ce qui me donne l'occasion de rappeler la nécessité d'ouvrir très rapidement le chantier sur le sujet, si ne voulons pas en rester au stade de l'incantation. Ils devront intégrer de nouveaux objectifs chiffrés sanctionnables, la mise en place d'indicateurs de résilience, tels le pourcentage de l'autonomie alimentaire territoriale, le développement des circuits alimentaires de proximité, les installations ou les conversions en vente directe, sans oublier le nécessaire accompagnement des agriculteurs dans la régénération des sols.

Les collectivités territoriales, elles aussi, ont de la volonté à revendre. Elles ont montré, ces dernières semaines, à quel point elles étaient essentielles pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Faire de nos EPCI des autorités organisatrices de l'alimentation durable et locale, et réunir tous les acteurs autour de la table pour prendre des décisions partagées et encouragées constitue une perspective à laquelle je vous sais très attaché. cette volonté, monsieur le ministre, est la vôtre, et que vous entendez consacrer énergie et moyens à la question de l'alimentation durable et locale. N'attendons pas pour repenser notre alimentation ! Il est désormais urgent de penser des systèmes alimentaires territorialisés.

Mon ancienne collègue Nelly Tocqueville, que je salue, et moi-même avons ces derniers mois travaillé sur ce sujet. Nous remettons l'ouvrage sur le métier et formulons des propositions que, j'en suis sûr, vous partagerez. Plusieurs choses me frappent : la qualité, l'envie et l'inventivité de tous les acteurs pour tendre vers une résilience alimentaire de qualité,

ma conception est claire : il faut assurer la santé nutritionnelle de nos concitoyens une alimentation de qualité, saine et durable, permise par nos agricultures partout sur le territoire.

équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé. Dans le

pour que les cuisines centrales puissent réaliser plus de 3 milliards annuels de repas à base de produits locaux, il devient absolument nécessaire de maîtriser la destination des terrains agricoles, lorsqu'ils sont libérés, et de pouvoir les attribuer aux cultures en déficit telles que le maraîchage ou les légumes de plein champ. L'alimentation collective nécessite en effet des cultures sur de grandes surfaces, afin de répondre aux besoins quantitatifs mais aussi parce que la massification de la production permet des prix plus bas, tout en laissant aux producteurs une marge suffisante.

des préemptions partielles pour les attribuer à d'autres fins agricoles, comme les cultures de plein champ. Enfin, il apparaît nécessaire, sur le plan de la gouvernance, de structurer et de renforcer les filières et les interfilières afin d'améliorer les questions de logistique, en faisant en sorte que tous les acteurs

Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous mettre en oeuvre pour que les conseils départementaux, au travers des PAT, soient les pilotes reconnus, légitimes et efficaces de l'organisation d'une production alimentaire locale et durable à destination des cuisines centrales ?

Dans mon territoire du Nord, sur la commune de Noordpeene en Flandres, un boulanger engagé montre la voie du circuit « ultracourt ». En juillet dernier, il a acheté un petit moulin autrichien pour moudre le blé d'une variété panifiable convenue avec avec l'agriculteur, cultivé sur la parcelle contiguë à sa boulangerie, et ainsi faire son pain. La farine obtenue préserve les oligoéléments et le gluten du blé, grâce à un procédé plus lent que dans le circuit industriel et une température ne dépassant jamais les 40 degrés : ça, c'est du pragmatisme ! Les produits pâtissiers sont, eux aussi, fabriqués grâce au lait acheté à un laitier de la commune. Les fruits proviennent d'un maraîcher voisin respectant la saisonnalité.

Le circuit « ultracourt » permet de recréer du lien et de développer une vie sociale parfois perdue dans certains de nos territoires. Ce nouveau dynamisme est un espoir pour nos communes. Mais si l'alimentation locale est autant plébiscitée actuellement, c'est parce qu'elle est synonyme d'impact carbone moindre. L'alimentation représente le quart de l'empreinte carbone des ménages français. Or ces derniers sont de plus en plus attentifs à leur impact sur l'environnement, notamment dans leur choix de consommation alimentaire. alimentaire. Votre ministère, avec le concours d'autres acteurs, a lancé au début du mois dernier un appel à candidatures pour expérimenter l'affichage environnemental des produits alimentaires. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre gaspillage et à l'économie circulaire. La Convention citoyenne pour le climat a aussi émis l'idée d'un « score carbone » sur tous les produits de consommation et les services. Quelles sont donc, monsieur le ministre, vos pistes de réflexion sur l'affichage du poids carbone de notre alimentation ? Je pense notamment à une définition, à un mode de calcul clair, et plus particulièrement à l'encouragement de ces pionniers parmi lesquels figure mon boulanger des Flandres.

de l'hôpital Lariboisière, qui met en lumière la présence de cadmium dans les engrais phosphatés, les pommes de terre et, en bout de chaîne, dans les urines humaines. Le cadmium est un métal lourd, classé comme « cancérigène certain » par le Centre

Que compte faire le Gouvernement pour préserver l'alimentation des Français de cette pollution au cadmium les engrais phosphatés ?

réplique. Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse. D'après les données dont nous disposons, les industriels sont en mesure de dépolluer les engrais phosphatés pour un surcoût évalué à seulement

Les recommandations alors établies traduisaient une ambition forte : bâtir une « chaîne alimentaire bénéfique pour les producteurs, les consommateurs, l'environnement et le climat », dans le cadre du pacte vert pour II a notamment été proposé de porter la part de l'agriculture biologique à 25 % des terres cultivées en Europe, à l'horizon 2030. D'autres propositions doivent être faites en lien avec la lutte contre le gaspillage alimentaire, ou concernant la nécessité d'un étiquetage nutritionnel, deux problématiques abordées au Sénat au cours de la session passée. En France, dans la continuité des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, qui a défini un objectif de 50 % de fermes en agroécologie pour 2040, le Gouvernement vient d'annoncer un plan de relance ambitieux pour l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est d'ailleurs ce qu'ont souligné plus de cent quarante acteurs de la transition agroécologique dans une tribune parue le 9 octobre dernier, en recommandant d'« accélérer la transformation de notre modèle agricole » et d'agir « pour une agriculture du vivant Se pose en même temps, et de manière accrue aujourd'hui, la question de notre indépendance protéique et de notre souveraineté, alors que la crise sanitaire a mis en exergue les effets désastreux pour les populations que pourrait avoir la rupture des circuits mondiaux.

Les sous-préfets de la relance interviendront-ils également sur ces sujets ? Les élus auront besoin de pouvoir identifier précisément les aides auxquelles ils peuvent prétendre lors de la mise en oeuvre de leurs propres feuilles de route. La

ce ne sera possible qu'avec une réelle volonté politique des territoires. Les PAT ont du mal à décoller. Pourtant, leurs enjeux sont nombreux : d'ordre économique, au travers de l'aménagement du territoire, de l'emploi non délocalisable, de l'installation ; d'ordre environnemental, avec la valorisation de nouveaux modes de production agroécologique ; d'ordre social, par l'éducation alimentaire, la création de liens, la valorisation du patrimoine. Monsieur le ministre, vous allez annoncer des moyens considérables pour les PAT. Pour autant, comment rendre plus efficient cet outil

du Gouvernement et encore moins celui du ministre de l'agriculture : c'est le plan de relance des Français, des agriculteurs et de ceux qu'ils nourrissent. Il nous faut donc absolument faire vivre toute cette famille. Les chambres d'agriculture jouent un rôle fondamental. C'est d'ailleurs pour

Notre groupe est un défenseur acharné et un fervent promoteur de l'agriculture paysanne, biologique, respectueuse de l'humain et de la planète, et rémunératrice pour le monde paysan.

En effet, le libre-échange détruit l'agriculture durable et locale en cassant nos normes. Il aggrave le réchauffement climatique en augmentant les émissions de gaz à effet de serre, avec des produits qui font parfois trois fois le tour de la planète ! Le meilleur exemple en est le CETA, ce traité de deuxième génération, ou traité mixte, signé entre l'Union européenne et le Canada, qui fait tomber les barrières tarifaires et douanières mais aussi les barrières non tarifaires, en s'attaquant aux normes sociales et environnementales ainsi qu'à nos services publics.

La crise sanitaire interroge de manière urgente notre autonomie et notre souveraineté alimentaires. La mondialisation crée des dépendances vitales malgré notre capacité à produire. Face à ce constat, comment envisagez-vous la nécessaire adaptation du Programme national pour l'alimentation (PNA) à l'éclairage de la crise actuelle ? Existe-t-il un nouveau plan Protéines végétales ? Ces sujets font-ils l'objet d'une réflexion partagée à l'échelle européenne ? Paradoxalement, vous semblez avoir abandonné le projet de loi foncière pour préserver les terres agricoles, facteur de lutte contre le changement climatique et de souveraineté alimentaire.

Vous allez consacrer une partie du plan de relance à ces objectifs. Les 80 millions d'euros dont vous avez parlé seront-ils également mobilisés pour accompagner la diversification des exploitations en circuit long vers les circuits courts, et pour permettre les nécessaires reconversions sociales et économiques ? les PAT pourraient être des obligations pertinentes pour engager les territoires en valorisant les subsidiarités, en organisant les besoins logistiques et les circuits de valorisation. L'intégration des PAT dans les SCOT et les Sraddet contribuerait à articuler ces politiques territoriales et faciliterait leur contractualisation. où en sont vos réflexions sur ces sujets particulièrement sensibles, qui méritent des réponses concrètes et factuelles ? La

ans que nos agriculteurs se battent face à la concurrence déloyale et aux hauts fonctionnaires de la Commission européenne, à Bruxelles. À force, ils s'épuisent et sombrent dans le désespoir : tous les deux jours, un agriculteur français se suicide. Nous étions autrefois l'un des plus grands pays agricoles du monde. Nous en sommes aujourd'hui réduits à consommer du boeuf aux hormones brésilien ou canadien, du poulet aux antibiotiques américain, du soja transgénique asiatique. Si nous voulons protéger nos agriculteurs et retrouver une alimentation durable, la première solution est de remettre des barrières douanières sur les produits que nos paysans produisent déjà. Nous devons partout favoriser les produits français, imposer au moins 70 % de repas locaux dans nos cantines. L'initiative de la commune de Châteauneuf-le-Rouge dans les Bouches-du-Rhône est à ce titre un exemple à suivre. des accords que des ministres, inconnus ou disparus, ont signés et de l'Union européenne, me direz-vous ? Sincèrement, je me moque de ces accords ! Un accord international rédigé par des bureaucrates et signé par des énarques ne vaut pas la vie d'un seul paysan français. Même s'il a reculé sur l'accord avec l'Amérique du Sud, ce gouvernement signe à tout-va les accords de libre-échange avec le Canada ou le Vietnam. Les paysans, ce gouvernement ne les comprendra jamais, car la paysannerie, c'est l'inverse de la Macronie : la paysannerie n'est pas en marche, elle n'est pas hors sol, elle a le corps et l'âme enracinés. On est paysan par amour et par passion, non pas pour « faire du blé », mais pour le faire pousser- nuance qui fait toute la différence ! La sachant fragile et précieuse, les paysans protègent la terre pour mieux la transmettre, en même temps qu'ils transmettent un savoir-faire et un art de vivre incomparables. Aujourd'hui, dans nos campagnes, nous entendons non pas mugir, mais mourir des hommes et des femmes qui nous font vivre. Pour une alimentation durable et locale, faisons nôtre cette déclaration de Guy de Maupassant à la terre française : « J'aime ce pays, et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines, ces profondes et délicates racines, qui attachent un homme à la terre où sont nés et morts ses aïeux, qui l'attachent à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même.

je n'ai pas arrêté de dire qu'il fallait inciter tous nos concitoyens à manger des produits frais et locaux. C'est ce qu'il y a de meilleur pour leur santé, pour l'environnement, pour nos agriculteurs et, souvent, pour leur portefeuille. Toutefois, vous vous trompez,

En 2010, l'excédent commercial agricole français était de l'ordre de 12 milliards d'euros. En septembre 2020, il n'est plus que de 3,98 milliards d'euros.

Madame la présidente, monsieur le ministre, la crise sanitaire et ses conséquences éclairent d'un jour nouveau le sujet de l'alimentation durable et locale. Nous sommes face à l'opportunité historique de réaliser pleinement la transition écologique de notre modèle agricole. En effet, si une telle transition est amorcée dans de nombreux domaines et dans plusieurs États membres, l'empreinte environnementale de notre alimentation reste importante. En mai dernier, l'Union européenne s'est dotée d'une stratégie, « De la ferme à la fourchette », qui ambitionne notamment de réduire de 50 % l'utilisation de pesticides chimiques, ou encore de disposer de 25 % de la superficie agricole en agriculture biologique d'ici à 2030. Pour atteindre ces objectifs ambitieux et nécessaires, nous devons relever ensemble plusieurs défis : la souveraineté alimentaire, la rémunération des producteurs, la capacité de nos concitoyens à acheter leurs produits et, bien entendu, le développement durable. Dans un récent ouvrage, Hubert Védrine explique que le concept de « compétitivité écologique » va s'imposer rapidement. Nous devons aujourd'hui tracer ce chemin. Monsieur le ministre, face à l'indispensable transition agroécologique, quelle position la France va-t-elle défendre dans le cadre des prochains grands rendez-vous européens, qu'il s'agisse de la réforme de la PAC, de l'adoption du budget européen ou encore de la stratégie « De la ferme à la fourchette » Pour la mise en oeuvre de cette stratégie, la Commission a prévu un calendrier réglementaire et législatif allant presque jusqu'en 2024. Ce calendrier vous paraît-il adapté ? La France souhaite-t-elle que l'examen de certains textes soit avancé ? La parole

Je vis dans un secteur de grandes cultures où les paysans sont pris dans une spirale infernale. Certains se sont réunis pour travailler la terre avec respect, cultiver du bio en circuits courts à portée de tous, en respectant les nappes phréatiques, mais surtout en donnant aux agriculteurs une rémunération honnête et un regard respectueux sur leur métier.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire sans précédent que nous traversons, et qui touche durement nos concitoyens, nous conduit irrémédiablement à interroger nos modes de consommation, en particulier la qualité de notre alimentation. De fait, la question alimentaire a pris une importance grandissante et elle est devenue aujourd'hui un nouvel enjeu de développement durable pour les territoires.

La problématique de l'agriculture de proximité, de la préservation du foncier et des activités agricoles est prioritaire. Vous le savez, la maîtrise foncière est l'un des principaux outils dont nous disposons pour permettre et encourager l'installation de nouveaux agriculteurs, en mobilisant du foncier ou en achetant en fonction des opportunités, en lien avec les Safer. Pourtant, alors même que le droit de préemption des Safer a été conforté par l'acquisition de la totalité des parts d'une société, il s'avère que de nombreuses acquisitions de terres agricoles par des sociétés parfois étrangères continuent de susciter interrogations et inquiétudes. Ainsi, les fonds de gestion, par le biais de sociétés, continuent d'acheter à des exploitants et à des prix parfois très élevés des milliers d'hectares dont les productions sont en règle générale destinées à l'exportation. Les mécanismes de contournement de notre législation mis en oeuvre par ces acheteurs, notamment la pratique des cessions partielles, démontrent clairement l'inefficacité de nos outils de régulation. Les conséquences de cette spéculation sont néfastes pour nos territoires, en particulier pour les nouveaux agriculteurs. Monsieur le ministre, ma question est donc simple : vous aviez annoncé en 2017 la préparation d'une grande loi foncière, qui devait être programmée d'ici à la fin du quinquennat. Quand proposerez-vous au Parlement ? Comment comptez-vous agir pour mieux réguler le foncier agricole et empêcher les contournements du droit de préemption des Safer ?

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous alimenter de façon saine et durable est devenu un enjeu majeur et constitue une véritable attente de la part de tous nos concitoyens. Des États généraux de l'alimentation en 2017 à la loi Égalim en 2018, l'ensemble des acteurs se sont prononcés. Ce sont autant d'enjeux sanitaires, écologiques, agricoles et économiques qui font la complexité du sujet. Une impulsion a été donnée par l'article 24 de la loi Égalim, qui prévoit que les repas servis en restauration collective publique, d'ici au 1 janvier 2022, devront compter au moins 50 % de produits alimentaires durables de qualité, dont 20 % issus de l'agriculture biologique. Nous souscrivons à cet objectif, mais nous sommes confrontés à des difficultés de mise en oeuvre parce que nous n'avons pas les moyens sur le terrain. Nous ne comptons pas assez de producteurs, pas assez de maraîchers Que l'on parle de souveraineté alimentaire ou d'alimentation saine et durable, les circuits courts devraient être notre objectif n° 1. C'est d'ailleurs une ambition tracée par le européen, avec la stratégie « De la ferme à l'assiette » présentée le 20 mai dernier par la Commission européenne. Pour atteindre l'objectif, il faut aider à l'installation de producteurs locaux et leur assurer des volumes et des prix rémunérateurs. Prévus par la loi d'avenir pour l'agriculture en 2014, quelque 190 projets alimentaires territoriaux (PAT) ont vu le jour. Le Gouvernement en voulait 500,

Par ailleurs, quelles positions défendra la France, dans le cadre de la réforme de la PAC, pour concilier la transition agroécologique et la prise en compte de la situation financière critique de nos agriculteurs ?

le travail de nos éleveurs fait notre fierté collective. Malheureusement, le confinement et les mesures de restriction appliquées à la restauration collective, aux restaurateurs ainsi qu'aux professionnels du tourisme renforcent aujourd'hui les difficultés que certaines filières animales connaissaient depuis plusieurs années. Je voudrais attirer particulièrement votre attention sur la situation des abattoirs de proximité, qui sont nombreux à rencontrer des difficultés en milieu rural.

du nombre de bêtes abattues : 1 200 aujourd'hui, contre 4 000 il y a quelques années. Le retrait de la société Arcadie au printemps a réduit son activité de moitié porté un coup fatal à cet abattoir, qui cumule 700 000 euros de dette, dont 200 000 euros de redevance due à la commune. Le maintien de ces abattoirs locaux est pourtant

et une économie circulaire conforme aux nouvelles attentes de nos concitoyens, pour maintenir aussi des emplois dans des territoires en difficulté. leur disparition entraînera le déséquilibre de nombreuses filières. Le label « veau élevé sous la mère », qui fait la fierté du Ribéracois, est aujourd'hui menacé. Monsieur le ministre, le volet « filières animales » du plan France relance a été doté d'une enveloppe de 250 millions d'euros, dont 130 millions d'euros spécifiquement dédiés à la modernisation des abattoirs et aux outils de première transformation. transformation. Que comptez-vous faire pour sauver nos abattoirs ruraux ? Quels leviers comptez-vous activer pour inciter les acteurs privés à investir dans ces structures essentielles à une alimentation durable et locale ?

M. Édouard Courtial. Monsieur le ministre, qu'il me soit d'abord permis de dédier cette question à la mémoire de Laurent Darras, agriculteur décédé à la suite d'un accident dans son exploitation, hier, à Villers-Saint-Frambourg-Ognon, dans l'Oise.

désertification vétérinaire, transmission des exploitations : la liste des défis auxquels ils sont confrontés est longue et en découragerait plus d'un. Vivre

Résultat, l'agriculture française décroche par rapport à ses concurrents. Pourtant, elle est un atout indéniable pour notre avenir, non seulement parce qu'elle assure notre souveraineté et notre sécurité alimentaire, et qu'elle est l'ADN de nos territoires ruraux, aussi parce qu'elle est un formidable moteur pour l'ensemble de notre économie et la vitrine d'un savoir-faire unique, reconnu et envié dans le monde entier. Nos agriculteurs sont les premiers écologistes. Ils respectent cette terre qu'ils ont su apprivoiser. Notre agriculture est sans doute l'une des plus durables, voire la plus durable, du monde. Elle atteint un niveau d'exigence inégalé, avec des produits de qualité dont nous pouvons être fiers.

le développement des circuits courts est une tendance émergente de la consommation alimentaire, largement confirmée depuis l'épidémie de la covid-19. Cette crise sanitaire a développé l'attrait des consommateurs pour les produits locaux et pour la traçabilité des aliments. Elle a également révélé le soutien et la solidarité des Français envers les producteurs de proximité. Une relation de confiance s'est construite ; il est indispensable qu'une politique de soutien économique et fiscale vienne pérenniser cette relation. Certes, ces filières bénéficient des aides de l'État, au même titre que les entreprises des secteurs touchés par la crise sanitaire. Cependant, au-delà des mesures d'urgence, nous devons conforter leur avenir. À ce titre, la loi Égalim n'a pas permis de mieux structurer l'offre alimentaire produite sur le sol français, comme le Sénat a pu le constater dans son bilan d'application de la loi. Elle n'a pas non plus apporté les bénéfices économiques attendus pour les agriculteurs locaux. En effet, leurs revenus restent insuffisants, alors que la demande pour leurs produits augmente et que des emplois pourraient être créés, si l'État soutenait ces filières de manière pérenne. Monsieur le ministre, vous avez évoqué au début de ce débat la signature d'une série d'engagements avec les supermarchés, pour favoriser l'agriculture de proximité.

Le débat qui nous réunit aujourd'hui, monsieur le ministre, vient opportunément mettre le sujet de l'alimentation durable, et donc celui de l'agriculture, au coeur de nos discussions. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Bien que cette thématique ne soit pas vraiment nouvelle, elle a pris ces derniers mois, à la faveur de la pandémie, un relief particulier. En effet, chaque Français a pu constater par lui-même, au fur et à mesure que les frontières fermaient, à quel point la souveraineté alimentaire de la France était nécessaire, à quel point le circuit court pouvait répondre aux besoins d'une population, à quel point la démultiplication des circuits d'achat devait faire l'objet de toute notre attention. À cet égard, la mise en place de maisons des producteurs au sein de plusieurs bassins de vie semble avoir apporté des réponses satisfaisantes, pour les consommateurs comme pour les agriculteurs. Le principe de ces structures est assez simple il s'agit de réunir des producteurs qui s'engagent à respecter une charte des bonnes pratiques garantissant la qualité de leurs produits, et de mettre à leur disposition des locaux ou du foncier pour qu'ils puissent vendre directement leurs produits de saison. Aujourd'hui, 37 départements participent à cette démarche et organisent plus de 2 500 marchés qui sont, en outre, devenus de véritables outils d'animation et de développement des territoires, tout au long de l'année. Néanmoins, si l'objectif est simple, la mise en oeuvre se heurte à deux difficultés majeures : le financement et la lisibilité. En ce qui concerne le financement, chaque création d'une nouvelle maison des producteurs est le fruit d'un partenariat entre les producteurs, la chambre d'agriculture et les collectivités locales.

Toutes les initiatives sont pertinentes, mais entre les plateformes des chambres consulaires, des associations d'élus, des collectivités, des commerces et des artisans de proximité, les professionnels et les consommateurs finissent par s'y perdre. Au sortir de la pandémie, face à des budgets contraints, nous verrons un élan réel pour mailler le territoire avec des structures nouvelles, qui mutualisent les forces de chacun. Les agriculteurs le souhaitent, les Français y souscrivent également. Vous savez combien les Français ont toujours manifesté un attachement historique et culturel à leur alimentation. Aussi, ma question est simple : quelle aide l'État serait-il prêt à à apporter pour la création de nouveaux marchés des producteurs ou la professionnalisation des marchés existants ? La parole

un formidable exemple de l'excellence française, mais un peu moins des autres marchés qui maillent notre territoire et ne sont pas souvent associés à certaines initiatives et politiques publiques que nous mettons en oeuvre.

Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Nous sommes tous unanimes, et vous le premier, monsieur le ministre, pour dire que l'accès à une alimentation saine, durable et locale est une priorité. d'une question autant de justice sociale que de santé publique, vous l'avez dit et répété. Notre débat a permis de mesurer combien les territoires sont essentiels au développement d'une alimentation de qualité et de proximité accessible à tous. Cet enjeu est au coeur du plan de relance et des mesures que vous avez pu, monsieur le ministre, tout au long de ce débat, exposer : création de circuits courts et lutte contre le gaspillage, pratiques exemplaires et filières locales. Il est évident que les territoires ont un rôle clé à jouer pour développer de véritables synergies alimentaires. Nos territoires ont un rôle clé d'assemblier à jouer, notamment sur la question de l'accélération de la transition agroécologique au service d'une alimentation saine, sûre, durable, locale et de qualité pour tous.

ce grand dessein que vous incarnez, lequel est l'alpha et l'oméga de votre action quotidienne, ne peut réussir que si l'on s'appuie- vous l'avez dit -sur la dynamique territoriale partagée par tous les acteurs.

Le renforcement des circuits de proximité doit être une priorité en vue, et ce n'est pas anodin, de redévelopper l'emploi dans les territoires et de réduire l'impact environnemental de notre alimentation.

Le sujet a été au coeur de nombre de programmes municipaux. Pour ne prendre que l'exemple du département du Nord, un grand nombre de communes et d'intercommunalités ont fait de l'alimentation durable et locale un véritable objet politique. Je ne compte plus le nombre d'élus délégués à l'alimentation durable et locale ; chacun pourra s'en féliciter.

L'accès de nos concitoyens les plus modestes, les plus isolés, à une alimentation locale saine, sûre, durable et de qualité est une priorité à laquelle nous devons consacrer tous les moyens financiers et toutes les énergies.